Je souhaite excuser l'absence de M. le président du Sénat, qui assiste aujourd'hui au congrès de l'Assemblée des départements de France. Je rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur le site internet du Sénat et sur Facebook. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun à observer, au cours de nos échanges, l'une de nos valeurs essentielles : le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole.

la colère gronde sur tout le territoire face à l'augmentation des prix du gaz, du fioul domestique et de l'essence. Cette colère est légitime, car elle exprime le sentiment d'assister à un véritable hold-up fiscal. Vous faites payer une fiscalité maquillée en vert aux familles populaires et aux classes moyennes. Or ce sont ces familles qui subissent déjà les salaires bloqués et la non-revalorisation du SMIC, et qui voient leurs pensions de retraite baisser avec la hausse de la CSG,

Alors que le réchauffement climatique entre dans un cycle infernal, vous trouvez le moyen de taxer le smicard qui gagne 1 153 euros et qui n'a d'autre choix que de faire 35 kilomètres par jour en voiture. Savez-vous, monsieur le ministre, qu'il y a aujourd'hui 18 millions de Français en zone blanche des transports publics ? Par contre, vous ne taxez surtout pas l'entreprise Total, qui réalisait, en 2017, plus de 8 milliards d'euros de bénéfices nets ! La lutte contre le réchauffement climatique est impérative ! Mais, pour la mener efficacement, arrêtez de fermer les petites gares ! Arrêtez vos bus « Macron », qui roulent au diesel ! Stoppez les activités de forage offshore de Total en Guyane ! Développez les transports publics, et parlons de la gratuité ! Taxez le kérosène et les croisiéristes ! Taxez Total et les sociétés d'autoroutes Mieux même : renationalisez ces dernières pour qu'elles contribuent à cet enjeu de société. Monsieur le ministre, allez-vous arrêter de taxer les Français et vous attaquer enfin aux lobbies

Oui, la fiscalité pèse sur ce prix, à hauteur de 3 à 7 centimes par litre de carburant. Nous avons pleinement conscience que cela crée des difficultés pour certains ménages modestes, et notamment pour ceux qui sont obligés de se rendre à leur travail en voiture, mais je voudrais dire deux choses. D'abord, nous assumons cette fiscalité ; elle est conforme à nos engagements pour le climat. Elle est conforme à notre lutte contre la pollution atmosphérique, qui tue des milliers de personnes chaque année. Nous préférons taxer la pollution plutôt que le travail. Et vous savez bien que les charges sociales et la taxe d'habitation des ménages ont baissé. Vous savez aussi que pour chaque euro de hausse de taxe sur les carburants, le Gouvernement rend,, 4 euros en baisse d'impôts ou de charges. Pour autant,

de se chauffer ou de se déplacer, les Français constatent que leurs factures augmentent dans des proportions insupportables. Les mécontentements montent de toutes parts dans le pays et, malgré les annonces, vous n'avez pas pris la mesure des difficultés que vivent nos concitoyens. Je pense à ceux dont les revenus sont modestes ou dont le pouvoir d'achat diminue, et qui sont à l'euro près pour boucler leur fin de mois. Je pense à ces ruraux qui sont captifs du carburant pour se déplacer ou se chauffer, à ces Français qui voudraient bien isoler leur maison pour payer moins cher leur chauffage. Le Gouvernement s'était engagé, par exemple, à transformer en prime le crédit d'impôt pour la transition énergétique. On attend toujours ; mais ce qui est sûr, c'est que les crédits correspondants sont divisés par deux dans le budget pour De surcroît, les Français se sentent grugés quand 20 % seulement des augmentations de taxes sont affectés à la transition. Ils ne voient pas où vous voulez mener le pays, quand il s'agit de faire face aux enjeux multiples et cruciaux de la transition énergétique et écologique. Ces enjeux, les Français les partagent ; cette transition, pour autant que les mesures prises soient justes et efficaces. Pourquoi, alors, les stigmatiser, les culpabiliser, les rendre responsables d'un état de fait qu'ils subissent entièrement et pour lequel vous ne proposez pas de réponse à la hauteur de leurs difficultés ? Monsieur le ministre, tout en engageant résolument la France dans la transition économique, sociale et environnementale, qui doit se faire au bénéfice de tous, quelles nouvelles mesures entendez-vous rapidement prendre pour répondre aux difficultés des Français ?

de transparence et de pédagogie s'agissant de l'utilisation des recettes fiscales prélevées au titre de la fiscalité écologique.

et Territoires. Le Président de la République a pris des engagements extrêmement clairs en matière de préservation du budget de la défense. Nous avons voté une loi de finances pour 2018 qui sanctuarise ce budget, et nous avons voté une loi de programmation militaire ambitieuse, qui augmente même les crédits de la défense, ce qui n'était pas arrivé depuis près de vingt ans. Les Indépendants ont salué cet effort.

qui devaient être prises en charge à hauteur de 50 % par la solidarité interministérielle, n'y seraient plus prises en charge que par le ministère de la défense. Ce n'est pas ce que nous avons voté. Ce n'est pas ce que nous avons soutenu. Et ce n'est pas possible Nous avons donc besoin d'éclaircissements sur ce point. À l'heure où le Président de la République est en itinérance mémorielle pour célébrer nos anciens combattants, ... où l'ensemble de la Nation salue la mémoire de nos combattants, à l'heure, surtout, où, à l'extérieur comme à l'intérieur, nos armées combattent pour défendre nos valeurs, il est important que nous puissions savoir où et comment vont être libérés les 404 millions d'euros qui manquent pour faire face à cette dépense nouvelle.

aux annulations de crédits du ministère de la défense, elles représentent moins de 1 % du budget dudit ministère. Elles n'auront aucune conséquence sur les commandes et livraisons de matériels au profit des armées,

seront intégralement respectés. Monsieur le secrétaire d'État, vous l'avez compris : nous sommes tout à fait capables de faire des économies sur d'autres missions ; mais, s'agissant de la défense, il faut que les engagements soient tenus : on ne doit rogner ni sur l'investissement, ni sur l'innovation, ni sur l'équipement des troupes.

Monsieur le ministre d'État, vous avez décidé d'augmenter une nouvelle fois la taxe sur les carburants ; vous assumez cette position de manière constante. Il est grand temps que vous preniez conscience de l'injustice qu'engendre votre politique, au lieu de vous contenter de mesures de circonstance en réaction à la colère des Français. Vous êtes le chef d'orchestre d'une fiscalité punitive, à défaut de dérouler la partition d'une écologie positive, unique clé d'une transition énergétique harmonieuse, capable d'emporter l'adhésion des Français. Cette politique confiscatoire est le point d'orgue de ce que vous essayez de vendre aux Français comme étant la symphonie du nouveau monde. Alors, monsieur le ministre, quelles nouvelles orientations décisives et stratégiques proposez-vous pour être à la hauteur des enjeux de la transition écologique que l'urgence climatique exige ?

Je veux souligner, monsieur le ministre, l'incohérence de votre politique de taxation énergétique, faite de volte-face permanentes. Soyons précis

vous prenez plus aux Français, mais donnez moins à la transition écologique. Le Président de la République affiche la volonté de taxer moins le travail et davantage le carburant. Mais le carburant permet aux Français d'aller au travail

les Pyrénées sont devenues une nouvelle route pour les populations migrantes : 50 000 personnes sont arrivées sur les côtes espagnoles depuis le début de l'année, ce qui représente la moitié des entrées sur le continent. Sa proximité avec la principale porte d'entrée européenne fait du Pays basque un lieu de transit important pour les migrants en provenance de Guinée, du Mali ou de Côte d'Ivoire : cent migrants arrivent tous les jours à Bayonne. La ville et la communauté d'agglomération font face à un vrai défi humanitaire : il faut mettre à l'abri avant l'entrée dans l'hiver ces populations fragilisées, constituées surtout d'hommes jeunes, de mineurs isolés, de femmes seules avec enfants. Elles peuvent compter sur de nombreuses associations, qui organisent l'aide aux arrivants et déploient un plan d'actions estimé à 55 000 euros par mois, mais la société civile ne peut pas tout. Monsieur le ministre, quel soutien l'État est-il en mesure d'apporter aux communes et aux intercommunalités pour répondre au défi humanitaire ? Quelles aides pour les départements de France qui prennent en charge les mineurs isolés ? Comment renforcer le contrôle aux frontières et lutter contre la prolifération des réseaux de passeurs ? L'Europe a progressé grâce au renforcement de l'agence FRONTEX et des actions extérieures ; mais, d'une part, pouvez-vous nous dire où en sont les négociations

de mobiliser une aide exceptionnelle de 140 millions d'euros à destination du Maroc, et j'ai échangé aujourd'hui même, à midi, avec mon homologue marocain pour faire en sorte que cette enveloppe permette de financer des opérations d'anticipation du risque migratoire.

Sur cette terre traditionnellement hospitalière qu'est le Pays basque, le populisme n'a pas sa place. La parole

À de multiples reprises, j'ai pu constater et regretter les difficultés parfois extrêmes vécues par les personnes en situation de handicap ainsi que par leurs familles dans l'organisation de leur vie quotidienne, face notamment aux démarches qu'elles doivent effectuer, qui sont complexes et répétitives. Lorsqu'il faut, par exemple, « redémontrer », à échéance régulière, le handicap de son enfant afin de bénéficier d'une continuité dans l'accompagnement, quelle souffrance et que de complications ! Quelle violence inutile ajoutée à des parcours de vie déjà très compliqués Le 19 juin dernier, Dominique Gillot, présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées, dont nous connaissons ici le travail, vous présentait des solutions concrètes afin de faciliter l'embauche et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Le comité interministériel du handicap, qui s'est réuni en octobre, avec l'ensemble des ministres, poursuivait le même objectif de simplification. À cette occasion, des annonces fortes ont été faites. Certains droits, comme celui d'avoir un accompagnant éducatif, seront attribués pour un cycle scolaire et non plus par année. Je pense aussi à la création d'un bonus « inclusion handicap » dans les crèches et à la majoration du complément de libre choix du mode de garde pour les assistantes maternelles, qui représentent des avancées. Dans le même sens, l'allocation d'éducation sera attribuée jusqu'aux vingt ans de l'enfant. Vous avez également évoqué l'attribution de droits à vie pour les personnes dont le handicap n'est malheureusement pas susceptible d'évoluer favorablement. C'est un progrès considérable ! Madame la ministre, alors que ces annonces vont donner lieu à des décrets, nous souhaiterions connaître le calendrier de mise en place de ces mesures très attendues par les personnes handicapées et par leurs familles.

citoyenneté des personnes handicapées sous tutelle. Je pense au droit de vote inaliénable et aux droits de se marier, de se pacser ou de divorcer sans recourir à l'autorisation judiciaire. Ces mesures sont discutées dans le cadre du projet de loi de réforme de la justice. Le Gouvernement a aussi souhaité avancer rapidement sur l'amélioration de l'accès au droit et sur la simplification des démarches. À partir du 1 janvier 2019, les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement verront leurs droits alloués à vie.

Les textes réglementaires seront publiés d'ici à la fin de l'année. L'ambition du Gouvernement se décline encore dans les budgets alloués au handicap, en hausse de 5 % en 2019- cet effort est inédit.

Sous l'effet, notamment, de la baisse des cotisations sociales sur les salaires et de la diminution de 30 % de la taxe d'habitation pour 80 % des foyers, l'INSEE prévoit une augmentation de 1,7 % du pouvoir d'achat au quatrième trimestre. Ces évolutions, certes fragiles, mais bien réelles, devraient redonner de l'optimisme aux Français. Et pourtant, le ressenti de beaucoup de nos concitoyens est tout autre : ils estiment que la hausse significative du prix des carburants et du fioul domestique- hausse de 15 % à 25 % suivant les produits -ampute fortement leur pouvoir d'achat. Ils en font porter la responsabilité aux taxes, donc au Gouvernement, alors que l'évolution du prix du pétrole brut représente 73 % à 82 % de cette hausse.

Face à l'émoi et à la contestation qui semble s'amplifier, le Président de la République assume et explique qu'il préfère taxer les carburants plutôt que le travail. On peut adhérer à ce concept, autant occulter le fait que la hausse du prix des carburants peut aussi amputer la rémunération du travail pour tous ceux qui, du fait de leurs horaires de travail, de leurs trajets ou de l'absence de transports en commun, sont obligés au quotidien d'utiliser leur véhicule pour travailler ou pour se rendre au travail. Cette situation est particulièrement fréquente- c'est même le cas général -dans les territoires ruraux. Comme l'envisage le Gouvernement, tous ceux qui sont fortement affectés par la hausse des carburants- notamment les salariés, mais aussi les travailleurs indépendants, les services et les soins à domicile, par exemple -doivent pouvoir bénéficier de mesures d'accompagnement. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous, au-delà des dispositifs liés à la transition écologique, nous apporter des précisions nous apporter des précisions sur la nature de ces mesures, leur financement et un calendrier de leur mise en oeuvre ? Veuillez conclure, mon cher collègue ! Enfin, la constitution d'un groupe de travail associant les parlementaires et ayant une mission de proposition, de suivi et d'évaluation de ces dispositifs d'accompagnement peut-elle être envisagée ?

Monsieur le Premier ministre, le vote qui a eu lieu dimanche dernier en Nouvelle-Calédonie a vu s'exprimer 81 % de nos compatriotes résidant

Je veux aussi associer à cet hommage Michel Rocard, qui a choisi, avec d'autres, la résolution non violente de ce conflit. Cela s'est traduit par trente années de paix et de dialogue.

que la poursuite du dialogue se fera dans le respect absolu des accords de Nouméa et de notre Constitution ? La parole

Elle a voté dans un calme et une sérénité qui ont été notés par tous. Que ce soient les 250 délégués qui veillaient au

n'est contesté par personne. C'est une excellente nouvelle, qui est due à l'engagement de l'ensemble des forces politiques de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au remarquable travail d'organisation réalisé à la fois par les services de l'État, par les maires et par l'ensemble de ceux qui se sont engagés et ont concouru à ce travail.

intervient au terme de trente années absolument exceptionnelles. Le processus engagé en 1988 par Michel Rocard, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, et poursuivi en 1998 sur l'initiative de Lionel Jospin,

a permis, en 1998, de modifier les conditions issues des accords de Matignon. S'il n'y avait pas ce consensus, il ne serait pas raisonnable de vouloir modifier ce cadre. Il faut savoir- je pense que nous pouvons nous accorder sur ce point, monsieur le sénateur -que si ce cadre a des avantages considérables- le respect de la paix civile, l'expression démocratique de la volonté des électeurs de Nouvelle-Calédonie -, il présente également- il faut bien reconnaître -un certain nombre, non pas d'inconvénients,

amplement -sur les transferts de compétences. Cette question a été instruite et travaillée par l'État avec les forces politiques.

la qualité de la discussion et l'émergence du consensus sont des conditions déterminantes du succès. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, il n'a pas été procédé en la matière, il est indispensable que le Gouvernement travaille avec l'ensemble des parlementaires et des forces politiques. C'est pourquoi je me tiens à la disposition de l'ensemble des groupes parlementaires pour faire régulièrement le point sur la question de la Nouvelle-Calédonie. La parole

Pas un jour ne passe sans que nos policiers et nos gendarmes soient caillassés, insultés et molestés. Leurs agressions se comptent par centaines et leur moral est au plus bas : ils ne se sentent pas soutenus, ils sont peu considérés et mal équipés. La vague de suicides se poursuit et s'amplifie, jusque dans des lieux hautement symboliques, comme un appel au secours. Le projet de loi de finances pour 2019 ne répond ni à leurs espoirs ni à leurs attentes. Il ne fait qu'entretenir une situation qui les a amenés là où ils sont. Pourtant, la violence ne cesse d'augmenter dans les villes comme dans les campagnes. Elle devient habituelle, voire permanente. L'insécurité gagne sans cesse du terrain. Les missions de nos forces de sécurité intérieure se multiplient constamment. La réponse pénale n'est pas en adéquation avec cette nouvelle forme de criminalité. La commission d'enquête sénatoriale sur l'état des forces de sécurité intérieure a travaillé pendant plus de six mois, mené près d'une centaine d'auditions, effectué de nombreux déplacements sur le terrain et rédigé trente-cinq propositions concrètes qui sont le reflet des attentes de ces hommes et de ces femmes qui nous protègent. Nos gendarmes et nos policiers attendent des réponses concrètes : il y va de leur sécurité et de celle de nos concitoyens. Monsieur le ministre, ma question est simple : dans votre plan d'action, quels moyens comptez-vous donner aux forces de sécurité intérieure pour stopper ce climat de violence qui s'accentue de jour en jour ? La

En deux ans, le budget du ministère de l'intérieur aura augmenté de plus d'un milliard d'euros. Dans quelques jours, je viendrai vous présenter un budget en augmentation de 3,5 %. Cela suffit-il pour régler tous les problèmes ? Non ! La réponse est non,

près de 4 500 postes dans nos écoles de formation, parce qu'il faut bien évidemment aussi remplacer les départs à la retraite, ce que nous ferons. Nous avons poussé au maximum les capacités de notre système

Madame la ministre chargée des affaires européennes, comment faire respecter la souveraineté française et la souveraineté européenne à la suite du retrait des États-Unis de l'accord par lequel l'Iran s'est engagé à geler son programme nucléaire ? Le retrait des États-Unis de l'accord de Vienne préoccupe notamment la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui estiment que le Moyen-Orient est plus stable avec cet accord que sans que le monde sera plus dangereux si le multilatéralisme est remplacé par le rapport de force dit bilatéral. Les États-Unis considèrent que leur politique étrangère doit être la nôtre. est l'effet de l'extraterritorialité des lois américaines et, en particulier, de la deuxième vague de sanctions qui s'appliquent depuis quatre jours à l'Iran, mais aussi à toutes les entreprises européennes. Aussi, madame la ministre,

comme vous l'avez relevé, le 5 novembre, les États-Unis ont rétabli l'intégralité de leurs sanctions contre l'Iran. Cette deuxième vague de rétablissement des sanctions vise les secteurs pétrolier et financier. La France regrette vivement la décision américaine. Nous l'avons dit publiquement, avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Haute Représentante de l'Union européenne. Ensemble, nous avons rappelé notre soutien à la préservation du, ou JCPOA, ainsi qu'à la défense de nos entreprises qui commercent légitimement avec l'Iran. À ce jour, l'Iran met en oeuvre ses engagements au titre de l'accord, comme l'a encore certifié l'Agence internationale de l'énergie atomique dans son dernier rapport. C'est la condition du soutien de la France et de ses partenaires et la raison pour laquelle les Européens, mais aussi la Chine et la Russie, sont déterminés à préserver l'accord et les bénéfices que l'Iran peut en retirer.

À court terme, le SPV vise à faciliter les transactions financières pour les entreprises qui souhaitent continuer de commercer avec l'Iran dans le respect du droit européen et international. À plus long terme, et au-delà du seul cas iranien, il s'agit de créer un outil de souveraineté économique pour l'Union européenne. Vous avez en effet parfaitement raison nous ne pouvons accepter que nos entreprises, quand elles respectent notre droit, soient les victimes de sanctions extraterritoriales. Je salue à cet égard, monsieur le sénateur, votre rapport d'information, qui s'inscrit dans ces orientations. Je vous sais mobilisé sur ces questions ; soyez assuré que c'est aussi ce que nous avons à l'esprit quand nous nous battons pour une Europe souveraine.

vous le savez tous, le Moyen-Orient est bien proche de l'Europe ; le pic de migration de 2015 nous l'a rappelé. C'est pourquoi tout ce qui peut être fait pour la stabilité du Moyen-Orient est positif pour nous autres Européens.

Nous pensions être définitivement libérés de ces pesticides neurotoxiques, qui sont redoutables pour les abeilles et l'ensemble de la biodiversité, mais aussi pour la santé humaine. nous apprenait hier qu'un recours auprès du Conseil d'État, porté par- j'ose le dire -l'abominable Union des industries de la protection des plantes menaçait le décret d'interdiction publié le 30 juillet 2018. Sur ce sujet, notre pays a pourtant audacieux et exemplaire. L'interdiction de ces produits avait été votée dès 2016, dans le cadre de la loi Biodiversité ; la récente loi dite ÉGALIM est venue renforcer cette interdiction en l'étendant aux molécules présentant le même mode d'action. Monsieur le ministre d'État, j'ai trois questions convergentes à vous poser. Pouvez-vous d'abord nous assurer que le Gouvernement mobilise tous les moyens dont il dispose pour défendre ce décret ? Ensuite, si le décret venait à être annulé, le Gouvernement s'engage-t-il à maintenir l'interdiction ? ? Des arrêtés de retrait des autorisations de mise sur le marché seront-ils pris, en particulier pour le thiaclopride et l'acétamipride,

pour porter politiquement cette interdiction et faire respecter une décision parlementaire correspondant aux attentes de nos concitoyens

mais aussi les agriculteurs, puisque la pollinisation constitue en quelque sorte un service rendu par les abeilles à la nature en général, mais aussi aux productions agricoles. Vous avez rappelé que la loi sur la biodiversité, qui a été adoptée en 2016, a permis

l'interdiction des néonicotinoïdes est et sera une réalité. D'ailleurs, ce référé suspension a été rejeté sur la forme ; sur le fond, il y aura bien sûr bientôt un jugement du Conseil d'État. La loi relative à l'agriculture et à l'alimentation a même élargi la liste des produits qui sont interdits à ce titre. Nous faisons activement valoir nos arguments en faveur de la validité de cette interdiction devant le Conseil d'État. La volonté du Gouvernement sur ce sujet est même confortée, comme en témoignent deux décisions récentes

soit copilotée par les ministres de l'agriculture et de l'environnement. C'est peut-être une demande de votre prédécesseur ; nous espérons vivement que vous la reprendrez avec force !

Les départements sont les collectivités de la solidarité, suffisamment proches pour être en contact avec les populations les plus déshéritées, suffisamment importantes pour assurer une solidarité entre les territoires.

Le coût du RSA et de l'APA augmente inexorablement. Sur ces deux seules allocations, le reste à charge pour les départements n'est plus supportable. Par ailleurs, il y avait 25 000 mineurs non accompagnés en 2017, ils seraient 40 000 en 2018. Or la contribution de l'État ne dépassera pas les 16 %. Comment s'étonner alors que les départements soient exsangues sur le plan financier ? Comment s'étonner que trente d'entre eux soient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations ?

Nous sommes loin du compte, très loin ! Monsieur le Premier ministre, madame la ministre, ma question est simple. Quel avenir voyez-vous pour les départements ? Ont-ils encore le droit d'exister à vos yeux ?

Madame la sénatrice, commençons par la fin, si vous voulez bien. Ah ! Il est vrai que les départements ont été parfois menacés dans leur existence,

Plusieurs actions vont être mises en place. Ainsi, dès 2019- ce n'est pas négligeable et c'était une demande forte des départements -, nous créerons un fichier national, qui permettra d'éviter de multiplier les procédures successives d'évaluation dans des départements différents. l'État assume pleinement sa mission régalienne. Les préfets pourront également procéder à des répartitions entre départements. Là encore, c'est une mesure pragmatique de nature à éviter des situations locales très tendues.

Je m'emploie, à la tête du ministère qui m'a été confié, à renouer le dialogue avec les départements. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller plus loin et, après en avoir discuté avec Dominique Bussereau au cours des trois dernières semaines, d'améliorer encore la prise en charge des mineurs non accompagnés, une fois qu'ils sont placés au sein de structures de l'aide sociale à l'enfance. Le Gouvernement a donc entendu ... Veuillez conclure, devant les présidents des conseils départementaux et j'espère que nos propositions seront tout autant entendues On a pourtant le sentiment, madame la ministre, que toutes les décisions prises tendent à étrangler les départements pour mieux les tuer. La dernière en date- et ce n'est pas la moindre ! -, c'est le rappel de plusieurs millions d'euros d'indus perçus au titre de la taxe d'aménagement, alors que la faute incombe à l'État.

-une barrière entre des arrondissements qui seraient devenus des carrés privilégiés et nos villes de banlieue, qui, encore une fois, seront mises au ban ? Madame la ministre, le transport, c'est la colonne vertébrale de la région d'Île-de-France.

Plutôt que de financer des infrastructures punitives et privatives en termes de pouvoir d'achat, ne pensez-vous pas que l'on devrait travailler sur ces problématiques de mobilité en concertation avec la région métropole dont c'est la compétence ?

pour remettre en état nos routes nationales, quand on prévoit un plan de désenclavement routier de 1 milliard d'euros, c'est bien parce que l'on est conscient que la voiture est importante pour se déplacer S'agissant des péages urbains, je voudrais mettre les points sur les i. Il n'est pas question que l'État incite quiconque à mettre en place des péages urbains, qu'il l'impose. Cette disposition existe dans la loi depuis près de dix ans et c'est d'ailleurs le Sénat, sur la base d'un amendement de votre ex-collègue Louis Nègre, qui l'a introduite en 2009 dans la loi Grenelle

: obligation serait faite de consulter les communes limitrophes en cas de mise en place d'un péage urbain et de fixer des tarifs plafonds. Je le répète : ce n'est pas l'État qui déciderait de mettre en place un tel outil et ce n'est pas non plus l'État qui en récupérerait les recettes. Ce sont les collectivités qui décideraient de le mettre en place si elles le souhaitent. Ce serait un outil parmi d'autres à leur disposition. C'est ce qu'elles nous ont demandé lors des Assises nationales de la mobilité.

Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement. Je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité au Gouvernement auront lieu mardi 13 novembre 2018, à seize heures quarante-cinq, et seront retransmises sur Public Sénat, le site internet du Sénat et sur Facebook.

Par cet amendement, nous souhaitons spécifier la nature du futur établissement public créé, l'agence nationale de la cohésion des territoires. Aux termes de ce texte, il s'agit d'une construction juridique sous forme hybride. Nous considérons pourtant que les missions confiées à cette structure doivent conduire à la définir comme un établissement public administratif. D'ailleurs, le Conseil d'État, dans son avis rendu à la demande du président du Sénat, a lui-même indiqué que « l'activité dominante de cette agence revêtira ainsi un caractère administratif ». Par ailleurs, et conformément aux doctrines du Conseil d'État en ce domaine, la nature des missions exercées et celle des ressources principales de l'établissement public constituent des critères en En l'occurrence, selon les propos du ministère, ces ressources seront principalement liées au budget de l'État, ce qui nous conduit à penser qu'il s'agira bien d'un établissement public administratif. Enfin, et par analogie en matière d'ingénierie publique et d'appui technique aux collectivités locales, le CEREMA est un établissement public administratif. N'est-ce pas la mission principale de cette agence que d'apporter de l'ingénierie et un appui technique aux collectivités ? Les formes des deux structures devraient donc être analogues, selon nous. L'ensemble de ces éléments nous conduit à préconiser que l'agence nationale de la cohésion des territoires

mais aussi qu'elle « peut être sollicitée par toutes les collectivités territoriales et leurs groupements ». Il s'agit de prévoir que les services de l'agence sont accessibles à toutes les collectivités, y compris aux communes, comme un guichet ouvert, pour reprendre l'engagement pris tout récemment par le Premier ministre. Cette agence sera destinée à apporter son soutien et son appui à tout le monde. Il faut que

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a souhaité maintenir, à l'article 5, la référence au département comme échelle première d'action de l'agence, dans un objectif de proximité : l'échelle départementale me semble la mieux calibrée pour répondre aux besoins des territoires, en particulier ruraux et périurbains.

de M. Morvan, sans qu'il faille nécessairement le préciser dans la loi. Au-delà, j'attire votre attention sur la modification apportée à l'article 5 par la commission

émettra un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Monsieur le sénateur, le Gouvernement entend la préoccupation exprimée par les auteurs de cet amendement quant au rôle et à la place de la région vis-à-vis de l'ANCT. En la matière, le Gouvernement tient à vous rassurer sur le fait que les régions ne sont absolument pas exclues de l'ANCT : elles ont au contraire pleinement leur rôle à jouer dans ce domaine, notamment au regard de leurs compétences en matière d'aménagement du territoire.

et faciliter les politiques d'intervention de l'État sur les territoires et réduire les inégalités qui nuisent à la cohésion et au développement équilibré des territoires. Nous proposons également que le Gouvernement s'engage dans l'élaboration d'une véritable stratégie nationale de cohésion des territoires, dans une démarche de coproduction de coproduction avec les élus. Cela nous semble très important. Cette stratégie permettrait de définir des objectifs de développement territorial et de réduction des inégalités, ainsi que les priorités nationales d'intervention de l'État. Elle pourrait également se décliner localement dans le cadre de contrats de cohésion territoriale signés avec l'État. Avec la création de cette agence, le Gouvernement revendique une approche nouvelle des relations entre l'État et les collectivités, pragmatique fondée sur les besoins exprimés sur le terrain. L'élaboration d'une stratégie nationale de cohésion des territoires et d'objectifs partagés avec des élus pourrait utilement consolider cette ambition. Quel est l'avis de la commission

par la rédaction du texte de la commission, qui précise que l'agence « assure la mise en oeuvre de la politique de l'État en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires et la coordination des interventions de l'État et des établissements publics ». Quant à la deuxième partie de l'amendement, faute de définir et d'apporter des précisions sur la stratégie nationale de cohésion des territoires et de prévoir la conclusion d'un contrat de cohésion territoriale à titre obligatoire, elle est dépourvue de caractère normatif. En revanche, je souhaite un engagement clair de la part du Gouvernement, madame la ministre, sur le vecteur juridique qui permettra de définir les contrats de cohésion territoriale, leur contenu et les objectifs qu'ils sont censés servir. Nous devons aussi avoir l'assurance que ce contrat va non pas simplement s'empiler sur les contrats existants, mais bien permettre de simplifier le paysage des instruments contractuels entre l'État et les collectivités territoriales. Je suis désolé, monsieur le président, d'émettre un avis défavorable

Mes chers collègues, il faudrait enfin réaliser que, une fois encore, le Gouvernement nous amuse

Il est clair que cette agence est un nouveau leurre destiné à faire patienter les élus, qui s'impatientent effectivement. C'est un moyen pour l'État de continuer à exercer sa tutelle sur les collectivités territoriales à moindre coût, en dégageant sa responsabilité et en donnant l'illusion d'un renforcement de l'autonomie des collectivités, et ce à moindre coût également. Vous aurez en effet remarqué que la charge financière de l'agence reposera sur l'État, les collectivités, sous forme de subventions ou d'achats de prestations,

Dans ce schéma, assurer l'équipement numérique du pays, la transition énergétique et, d'une manière générale, les équipements publics d'intérêt national et le service public relève de la responsabilité non plus de l'État, mais des collectivités, lesquelles auront la chance insigne d'être soutenues par l'agence

outre que les attributions concernant les infrastructures n'étaient pas précisées ? On craignait en effet que Julien Denormandie, qui assumait avec succès cette mission jusqu'alors, en soit dépossédé.

dit, j'ai bien compris que ce point posait certaines difficultés aux porteurs du texte, mais aussi à votre ministère, dans un souci d'efficacité, mais également de recherche de consensus, et après avoir longuement évoqué cette question avec l'ensemble des acteurs, je me rallierai aux amendements visant à conforter cette intégration immédiate, sous réserve

précisé que l'exercice des missions de l'agence ne peut se concevoir sans une articulation étroite entre les différents niveaux de collectivités,

du soutien et de l'expertise de l'agence nationale de la cohésion des territoires, y compris en amont de la construction des projets. À défaut, cette agence passera totalement à côté de son rôle de soutien logistique, technique et financier aux collectivités qui en ont le plus besoin.

a fait l'objet d'une mesure préventive d'évacuation il y a un an. Le département a pris seul en charge la construction d'un équipement provisoire à hauteur de 12 millions d'euros.

à la construction de bâtiments publics, de commerces et d'habitations. Ainsi, un certain nombre de collectivités territoriales voient leurs projets d'aménagement et de construction bloqués en raison du coût des études et des travaux induits par la dépollution des sols. Nous proposons donc que l'agence nationale de la cohésion des territoires permette aux collectivités territoriales, mais aussi aux aménageurs publics, de bénéficier de l'ingénierie et de l'action territoriale de l'État et de ses opérateurs en matière de dépollution des sols. C'est

: La parole est à M. Patrice Joly. Dans la rédaction issue des travaux de la commission, l'agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission de soutenir les projets locaux en faveur du maintien des services publics, de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, de la transition écologique, de la lutte contre le changement climatique, de l'accès aux soins et du numérique. Il est proposé de compléter cette liste par l'accès aux transports. La mobilité, on le sait, est un enjeu indispensable à la cohésion sociale, à la dynamique de l'emploi et à l'accès aux services dans tous les territoires. Il convient donc de répondre prioritairement à ces besoins de mobilité du quotidien en veillant à un aménagement du territoire équilibré. L'amendement

l'idée d'un opérateur de rattrapage des équipements qui permette de mobiliser les financements et les ressources de l'État. Pour répondre à cette ambition, notre amendement propose de concentrer les efforts de l'État au profit des territoires nécessitant un accompagnement prioritaire. Il nous semble donc que l'offre d'ingénierie de l'État doit prioritairement se tourner vers les territoires en difficulté, d'autant que de nombreux départements sont déjà organisés pour mettre en place un appui local et n'auront pas recours aux services de l'agence. Par ailleurs, l'agence doit répondre aux attentes de simplification et de transparence sur l'ensemble des dispositifs qui peuvent être mobilisés par les acteurs locaux. Pour répondre à ce besoin de lisibilité, il pourrait être envisagé une plateforme de recensement de l'ensemble des dispositifs dédiés à la cohésion et à la solidarité des territoires, qu'il s'agisse d'ingénierie ou de financements mobilisables par les porteurs de projets. Notre amendement vise ainsi à organiser les missions de l'agence autour de trois orientations : premièrement, une mission générale d'accompagnement des territoires ; deuxièmement, une simplification des dispositifs d'aide et une plus grande transparence troisièmement, une intervention renforcée auprès des territoires les plus en difficulté. Ce recalage des missions permettra à l'agence d'intervenir prioritairement en faveur des territoires les plus démunis et les plus défavorisés. L'amendement

en mobilisant et en coordonnant les moyens en ingénierie et en financements au profit des collectivités territoriales, et ce pour donner davantage de lisibilité et d'efficacité à l'intervention de l'État dans les territoires. Jusqu'à maintenant, le développement de l'ingénierie publique s'est opéré de manière peu cohérente, générant un manque de lisibilité entre les différents acteurs. Cette situation comporte également un risque

Afin de remédier à cette situation, l'agence pourra développer son offre d'ingénierie, dans le cas où serait observée de manière objective une carence de l'offre privée dans les territoires. Cet amendement permettrait ainsi d'articuler harmonieusement les différentes offres qui peuvent exister en matière d'ingénierie territoriale.

et parapublique : les agences techniques départementales, les sociétés publiques locales, les syndicats mixtes, etc. Il paraît donc extrêmement urgent d'organiser une ingénierie territoriale performante,

En effet, nous estimons que la définition actuelle est lacunaire et ne permet pas de distinguer ce qui relève de la compétence régalienne de l'État et ce qui peut être externalisé au sein d'une agence, opérateur de l'État. À défaut de précision, c'est ainsi la compétence de l'État en matière d'aménagement et de cohésion des territoires qui serait transférée à la future agence, ce qui n'est évidemment pas souhaitable, puisque nous craignons que cette externalisation ne rime une nouvelle fois avec désengagement et déresponsabilisation de l'État. Nous estimons ainsi, et même s'il est précisé que le rôle de l'agence est celui de la mise en oeuvre, qu'il convient de bien préciser que l'État conserve une compétence à titre principal en matière d'aménagement du territoire. La politique nationale ne peut en effet se résumer à une approche de guichet et donc à l'addition de prestations clients, comme le suggère le rapport Morvan. Il s'agit par ailleurs de mieux définir les compétences de l'agence aux côtés des représentations territoriales des autres opérateurs de l'État, tels que l'ANRU, l'ANAH, le CEREMA, ou encore l'ADEME, mais également des services déconcentrés de l'État. À nos yeux, l'intervention de l'agence n'épuise pas la compétence de l'État et se place en complémentarité. Enfin, et par conséquent, les auteurs de cet amendement considèrent que la mission de l'ANCT, la réelle plus-value de cette agence au titre de l'aménagement du territoire, doit être principalement celle d'accompagner les territoires dans leurs projets locaux, notamment la conception, réalisation et la mise en oeuvre de leurs documents d'urbanisme que sont les schémas régionaux climat air énergie, les plans climat air énergie territoriaux, les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les SRADDET, les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, et les plans locaux d'urbanisme, les

du préfet. L'article 2 de la proposition de loi, qui précise les missions de l'agence nationale de la cohésion des territoires, a fait l'objet de compléments de la part de la commission qui s'avèrent utiles et bienvenus pour clarifier le rôle et les missions de l'agence. parmi ces ajouts figure une mention selon laquelle l'ANCT aurait notamment pour mission d'assurer « la coordination des interventions de l'État et des établissements publics » en matière d'aménagement du territoire. Si l'ANCT constitue une simplification dans la mobilisation des opérateurs de l'État, elle n'a cependant pas vocation à se substituer au pouvoir du représentant de l'État dans les territoires.

des compétences du préfet. C'est une compétence propre. Il ne faut donc pas confondre les compétences propres du préfet, d'une manière générale, et celles de son rôle de représentant de l'ANCT sur les territoires. Donc, il ne s'agit nullement de remettre en cause ou d'amoindrir le rôle de l'agence, mais simplement de bien qualifier la « double casquette » du préfet.

Cet amendement vise à préciser que l'agence nationale de la cohésion des territoires pourrait être consultée sur l'impact des politiques publiques et des projets de lois

qui n'est absolument pas traitée par cette proposition de loi. Pourtant, l'on nous dit que le commissariat général à l'égalité des territoires sera demain, sauf son pôle régalien, totalement absorbé par l'Agence. Or, parmi les missions principales de ce commissariat général à l'égalité des territoires, aujourd'hui, figure bien la définition et la mise en oeuvre de la politique de la ville. Nous nous permettons à cette occasion de faire un bref retour en arrière. Il faut savoir que le commissariat général à l'égalité des territoires résulte de la fusion de trois entités la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, mais également le secrétariat général du comité interministériel des villes et l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Un pan très important des missions de cette structure correspond donc à l'élaboration de la politique de la ville. Or, à aucun moment, il n'est fait mention de ces compétences pour l'ANCT. La question est donc la suivante, madame la ministre : est-ce à dire que celles-ci disparaissent ? Et je ne doute pas de la véracité de votre réponse. Mes chers collègues, j'ai été interpellé par de nombreux élus de ces quartiers. Ils sont très inquiets de ces évolutions, et ce d'autant plus que le plan Borloo, tant attendu, est tombé dans un grand trou noir. noir. Nous proposons donc de reprendre pour la définition des missions de l'agence le contenu du décret qui définit les compétences du commissariat général à l'égalité des territoires en matière de politique de la ville. Nous demandons que l'agence nationale de la cohésion des territoires mette en oeuvre la politique nationale d'égalité des territoires et qu'elle soit chargée, en particulier, de la mise en oeuvre de la politique de la ville. Il ne s'agit pas de définir cette politique, puisque c'est une prérogative qui appartient à l'État, mais bien de s'assurer que l'ANCT soit la cheville ouvrière de sa mise en oeuvre aux côtés de l'ANRU, qui sera liée également à cette agence. Enfin, de manière pratique, nous estimons que cette définition complétée des missions de l'agence permettrait de sécuriser celle-ci juridiquement. En effet, une telle définition permettrait de respecter le principe de spécialité qui ordonne une définition précise et complète des missions du nouvel établissement public.

le texte actuel de la proposition de loi fait référence aux collectivités territoriales dans leur ensemble. Comme nous l'avons dit à l'article 1, les communes font donc naturellement partie du public cible de l'agence.

défavorable. L'amendement n° 50 rectifié inclut dans les missions de l'agence la fourniture d'un soutien aux entreprises et développeurs dans plusieurs domaines. Néanmoins, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable souhaite que l'agence s'adresse en priorité

par l'amendement de notre collègue Loïc Hervé à l'article 1. En outre, plusieurs éléments ne relèvent pas du domaine de la loi : il en va ainsi de la plateforme de contenus mentionnée au premier alinéa de son dispositif, ainsi que de la mission de veille et d'alerte territoriale, qui constituent des activités purement opérationnelles et administratives. La commission émet donc un avis défavorable. S'agissant

Au-delà, un rappel me semble important : les personnes publiques ont bien le droit d'intervenir sur un marché économique, à condition de justifier d'un intérêt public. Il résulte d'une jurisprudence administrative constante que, lorsqu'une personne publique intervient sur un marché, elle doit le faire dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie et présenter un motif d'intérêt général justifiant cette intervention. Au nombre de ces motifs figurent, par exemple, l'insuffisance, la carence ou l'inexistence de l'initiative privée, de même que l'économie réalisée grâce à cette intervention. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter sur ce point et cet amendement procède à une clarification utile. La commission émet un avis favorable. En ce qui

de M. Gontard, votre rapporteur vous propose de vous en tenir à la rédaction adoptée par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour des motifs de clarté du droit. ailleurs, il convient de bien faire apparaître la mission de coordination des interventions de l'État et de ses établissements publics, qui serait supprimée en cas d'adoption du présent amendement, alors qu'elle est essentielle pour permettre à l'agence d'être pleinement efficace dans les territoires.

pivot en matière de coordination des interventions de l'État, ainsi que le précise le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, mais la spécificité de l'ANCT est précisément sa vocation à incarner un guichet unique au bénéfice des collectivités territoriales, pour les actions entreprises par l'État et ses établissements publics, au premier rang desquels, en l'espèce, l'ADEME, l'ANRU, le CEREMA et l'ANAH. La commission émet donc un avis défavorable. L'amendement n° 6 rectifié est intéressant, car il vise à inciter à une plus grande prudence dans la conception des lois et règlements au regard de leurs éventuelles et réelles conséquences pour l'aménagement des territoires. Néanmoins, il pose une difficulté on imagine mal un établissement public rattaché à l'État et sur lequel un ministre, quel qu'il soit, exerce une tutelle se prononcer sur l'opportunité et le contenu des politiques publiques en matière d'aménagement du territoire. Dès lors, il conviendrait plutôt d'inclure un volet dédié à l'aménagement du territoire dans les études d'impact assorties aux projets de loi. Cette idée se rapproche d'ailleurs de celle exprimée dans le remarquable rapport. Pour toutes ces raisons, la

au regard de la rédaction actuelle de l'article 2, qui identifie bien des éléments de la politique de la ville dans le champ d'action de l'agence. La mention du développement de la participation citoyenne est peu précise. Le fait que l'agence assure l'évaluation des politiques publiques en matière d'égalité des territoires ressort de la compétence d'une direction d'administration centrale, à l'image du CGET. Ce n'est en revanche pas le rôle d'un établissement public, qui doit assurer la mise en oeuvre d'une politique publique. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

L'amendement n° 61 de M. Dantec fait l'objet d'une demande de retrait. Il a pour vocation de préciser que l'ANCT aura un rôle de diffusion des bonnes pratiques, ce qui sera satisfait sans qu'il soit besoin d'inscrire une telle disposition dans la loi, car cela relève de la mission de tout opérateur. Concernant

une mission de recensement et de publication des dispositifs locaux, nationaux et européens susceptibles d'être mobilisés en faveur de l'aménagement du territoire.

Je tiens à rappeler que la préparation des projets de loi et des décrets est une compétence de l'État, qu'il exerce au travers de ses services d'administration centrale. De son côté, l'agence est un opérateur de l'État, et il ne relève pas de la mission d'un opérateur, quel qu'il soit, d'apprécier les projets de loi

il me semble essentiel de ne pas chercher à circonscrire le périmètre géographique d'intervention de l'agence, car cette dernière, pour être véritablement au service de tous les territoires et de toutes les collectivités, doit pouvoir intervenir dans tous les domaines. C'est la raison pour laquelle je demande le retrait

Notre collègue Savoldelli y est certainement allé un peu fort. Toute la question est effectivement de savoir si la dépollution des sols, dans les exemples que nous avons donnés en termes d'aménagement, peut être comprise dans la transition écologique. Nous avons un doute. Donc, nous préférerions que cela soit inscrit

en première couronne parisienne, mais aussi dans les territoires au passé industriel important, qui connaissent ce type de difficultés. Les élus locaux que nous avons été ou que nous sommes encore, mais avec des responsabilités autres, savent que la question est extrêmement difficile à traiter et que, sans soutien de l'État, on n'y arrive pas.

explication de vote. Pour abonder dans le sens de mes collègues, je dirai que la question de la pollution et de la dépollution des sols est probablement ce qu'il y a de plus vertueux en termes d'écologie, puisqu'il s'agit de reconstruire la ville sur elle-même et sur des secteurs qui, jusqu'à présent, avaient été déconsidérés,

d'infrastructures, de climat et d'énergie, intervient régulièrement sur le sujet de la pollution des sols. Cela irait donc mieux en l'écrivant, d'une certaine façon. La mesure ne coûterait absolument rien,

on ne dit que l'agence a un rôle de capitalisation de ce qui remonte des territoires, pour en faire un élément fort de sa stratégie, y compris pour formuler des propositions à d'autres territoires ayant des problématiques similaires. J'entends bien, madame la ministre, qu'une loi ne doit pas être bavarde. Mais il faudrait donner à l'État ce rôle

En ce qui concerne la configuration de l'agence, l'article 2 de la proposition de loi définit les missions qui seront les siennes et intègre, à ce titre,

Pour l'instant, je le disais ce matin, aucune analyse ne démontre la pertinence de fusionner tous ces opérateurs, pas plus que les raisons qui ont conduit le Gouvernement à retenir l'EPARECA et l'Agence du numérique de préférence aux autres opérateurs intervenant au profit des territoires.

pas suffisamment éclairés pour pouvoir légiférer utilement. S'agissant plus particulièrement de l'Agence du numérique, faut-il le rappeler, elle pilote le plan France très haut débit, donc l'un des chantiers actuels les plus structurants de l'aménagement du territoire, avec des objectifs très

est à Mme la ministre. L'objet de cet amendement est de préciser que les syndicats mixtes ouverts peuvent également, comme les syndicats mixtes fermés, donner leur accord pour des opérations relevant du champ de compétence de l'EPARECA.

des établissements dont l'accord doit être préalablement requis. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité supprimer la référence du CGCT relative aux syndicats mixtes fermés, pour ne pas exclure les syndicats mixtes ouverts.

Comme nous l'avons déjà exposé lors de la discussion générale, notre groupe estime que l'intégration de l'Agence du numérique, dès la création de l'ANCT, est une condition de la réussite de cette dernière. On ne peut pas, d'un côté, reprocher la création d'une énième structure administrative et, de l'autre, ne pas donner à l'ANCT les moyens de ses ambitions, en la vidant d'une partie essentielle de ses missions. Or le numérique est un levier fondamental du développement économique des territoires et de la modernisation des services publics. Comme l'énonce le Conseil d'État dans son avis, ce nouvel établissement public « regroupera trois des structures pouvant intervenir au profit des collectivités territoriales, notamment l'Agence du numérique, qui joue un rôle essentiel dans la réduction de la " fracture numérique ", et restreindra ainsi le nombre de leurs interlocuteurs ». À notre sens, le report à 2021 de l'intégration de l'Agence du numérique est doublement un facteur de déstabilisation pour cette agence elle-même, puisqu'elle sera davantage préoccupée par l'achèvement du plan France très haut débit pour 2022- il répond à un besoin essentiel, au demeurant - ; pour l'ANCT ensuite, qui doit pouvoir exercer le plus rapidement possible les missions qui vont lui être dévolues pour répondre aux besoins des territoires. Or elle aura déjà, en 2021, finalisé la fusion du CGET et de l'EPARECA. Comment, dès lors, s'assurer de la cohérence de l'organisation de l'ANCT et de la coordination des services et opérateurs de l'État ? Tout simplement, si l'on peut dire, en organisant dès le départ la fusion des trois opérateurs ! Pour tout dire, nous craignons que, à terme, l'intégration de l'Agence du numérique ne soit tout simplement abandonnée. C'est pourquoi nous souhaitons supprimer ce report. Nous nous félicitons, au passage, que les positions des uns et des autres aient évolué ces derniers jours pour parvenir à une solution qui profitera en premier lieu aux collectivités territoriales. Nous tenons également à préciser un point, pour que le débat ne souffre d'aucune ambiguïté : il n'est absolument pas question pour nous d'intégrer à l'ANCT la French Tech. Il va de soi que la French Tech n'a pas vocation, par sa nature, à se fondre dans un établissement public qui travaillera pour les collectivités territoriales. Elle restera donc adossée au ministère de l'économie et des finances, afin qu'elle puisse poursuivre sa mission de promotion des entreprises françaises à l'international.

un arbre de plus dans la forêt des établissements publics de l'État, il convient de maintenir l'intégration de ces deux structures, dont les missions sont essentielles à la cohésion des territoires. J'émets donc un avis défavorable. La commission est en

Au-delà, il semble peu réaliste d'assigner cette mission à l'agence, car la mobilité des ménages est déterminée par de très nombreux facteurs allant au-delà de la volonté politique. En revanche, cet amendement pourrait être satisfait

à intervenir pour maîtriser et favoriser les flux de population. Une telle mission me semble très éloignée de son objet.

c'est un véritable enjeu que de gagner le pari de la reconquête démographique. On l'a dit, la population de la France va augmenter de 10 millions d'habitants dans les trente prochaines années. Si, dans les territoires ruraux, l'agence n'a pas pour mission d'accompagner les politiques d'accueil de nouveaux habitants menées par les collectivités,

à M. Jean-Jacques Lozach. L'agence nationale de la cohésion des territoires doit permettre de mutualiser un certain nombre de moyens et de ressources et d'alimenter au niveau national un corpus méthodologique et politique, notamment dans le domaine du développement territorial intégré. Elle doit être un média qui rapproche l'offre et la demande en matière d'installation, de transmission ou de reprise. La création d'une plateforme dédiée permettra de favoriser les volets d'ingénierie, d'expérimentation, de formation, de centre de ressources, de conseil et la dimension opérationnelle que l'État lui confiera.

de l'aménagement du territoire et du développement durable. En outre, la mention d'une plateforme de mise à disposition de données, de même que la précision inscrite au second alinéa concernant

l'agence. Nous nous réjouissons que la commission ait rejeté l'amendement du rapporteur, qui tendait à transformer ce conseil d'administration en un conseil de surveillance. Nous nous réjouissons également que l'État, contrairement au texte initial, ne soit plus majoritaire au sein de ce conseil. Pour autant, nous continuons de vouloir faire évoluer cette représentation. Nous considérons qu'il convient de donner une place prépondérante, c'est-à-dire majoritaire, au groupe des représentants des collectivités, des parlementaires et des représentants des personnels, afin de faire de cette agence un réel outil au service des collectivités territoriales. Une telle définition permettrait d'initier un changement majeur dans les rapports entre l'État et les collectivités, marqués depuis des décennies par la verticalité du pouvoir. Comprenons-nous bien : nous ne voulons pas que l'agence devienne un outil de recentralisation, mais qu'elle inaugure de nouvelles formes de coopération et de dialogue permettant aux collectivités d'être mieux entendues et mieux respectées. Ce signe est attendu, notamment après des mois marqués par un mépris gouvernemental, qui s'est traduit par une désertion des associations d'élus de la table des discussions. Nous ne pouvons pas en rester là, et nous souhaitons donc que ce texte envoie des signes tangibles d'une vision renouvelée d'une décentralisation qui ne rimerait ni avec désengagement ni avec autoritarisme. Enfin, nous souhaitons affiner la représentation des collectivités afin de permettre une représentation de tous les échelons territoriaux et de toutes les réalités territoriales, à la fois urbaines et rurales. Parmi les représentants des collectivités territoriales, nous proposons donc que soient nommés au moins un représentant sur proposition de l'Association des maires de France, un représentant sur proposition de l'Association des maires Ville et banlieue de France, un représentant sur proposition de l'Association des maires ruraux de France, un représentant sur proposition de l'Association nationale des élus de montagne, un représentant sur proposition de l'Assemblée des communautés

madame la ministre, pouvez-vous nous préciser pourquoi les représentants des personnels sont comptabilisés dans le collège des élus, alors qu'ils travaillent dans l'établissement

Lors de cette réunion, les représentants de l'État nous ont dit qu'ils étaient membres de plein droit de la commission, mais qu'ils ne pouvaient pas prendre part au vote.

la proposition qui est faite de donner un réel poids au collège des élus locaux semble de bon sens. Dans ses grands mouvements, la décentralisation

La composition du conseil administration de l'agence nationale de la cohésion des territoires doit en effet permettre une large représentation des représentants des collectivités, puisque c'est une

même si l'agence intervient au profit des territoires, et donc de leurs élus, je rappelle qu'il s'agit d'une agence de l'État, dont les moyens d'intervention, qu'ils soient financiers ou techniques, sont des moyens de l'État.

5,2 milliards d'euros en fonds propres que la Caisse des dépôts et consignations consacrera à la politique d'aménagement du territoire d'ici à 2022, en plus des prêts qui pourront être mobilisés. Au regard de l'importance des financements qu'elle apporte, mais aussi de son expertise reconnue en matière d'accompagnement des projets portés par les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, qui dispose d'un statut juridique particulier, doit être représentée au sein du conseil d'administration de l'agence nationale de la cohésion des territoires.

Les territoires ultramarins connaissent des enjeux spécifiques en termes d'aménagement du territoire au regard de leurs contraintes géographiques- nous pensons aux enjeux en termes de mobilité, d'indépendance énergétique, de logements, d'urbanisme ou encore de prise en compte des risques naturels. Dans la logique de la proposition de loi, qui souhaite partir des besoins exprimés par les territoires, le présent amendement vise à garantir la représentation des territoires d'outre-mer au sein du conseil d'administration de l'agence, en introduisant un représentant ultramarin parmi les représentants des collectivités territoriales,

pour présenter l'amendement n° 49. Les entreprises d'ingénierie privées de proximité constituent des acteurs essentiels engagés au niveau local, qui mettent leur expertise et les solutions qu'elles développent à disposition des collectivités territoriales et des populations. collectivités territoriales et des populations. Ce sont ainsi près de 21 000 entreprises employant 220 500 collaborateurs qui interviennent auprès des collectivités dans la définition, l'accompagnement et la mise en oeuvre de leurs projets de développement. La présence de représentants des acteurs de l'ingénierie privée dans les instances de l'agence est une condition essentielle de réussite de la mobilisation générale en faveur des territoires. Elle s'inscrit dans la volonté du législateur de doter l'agence d'une organisation et d'un fonctionnement innovant et efficace. Le présent amendement vise donc à garantir un dialogue permanent entre les différents acteurs, en intégrant des personnalités qualifiées représentatives du secteur de l'ingénierie privée au conseil d'administration de l'agence nationale de la cohésion des territoires. Il s'agit ainsi d'assurer une cohérence de l'offre d'ingénierie publique et privée sur tous les territoires.

a pour objet de rétablir une prédominance de l'État au conseil d'administration de l'agence. Il ne s'inscrit pas dans la logique de la rédaction adoptée par la commission, qui vise à instaurer la parité entre l'État et les collectivités au sein du conseil d'administration. L'avis est donc défavorable.

rééquilibrer le conseil d'administration en faveur des élus locaux et nationaux. La parité étant un souhait exprimé par la commission, c'est naturellement un avis favorable.

pose toujours une difficulté d'ordre juridique et pratique, car il tend à ériger les deux députés, les deux sénateurs et les représentants du personnel en arbitre, au sein du conseil d'administration, face à l'État,

à la demande du président du Sénat, la précision selon laquelle les représentants de l'ANRU, de l'ANAH, de l'ADEME et du CEREMA assistent au conseil d'administration de l'agence relève du domaine réglementaire. Ensuite la volonté de la commission est d'instaurer la parité, comme je l'ai déjà dit, entre les représentants de l'État, de ses établissements publics, ainsi que les personnels de l'agence, d'une part, et les représentants des collectivités territoriales et du Parlement, d'autre part.

l'amendement n° 23 rectifié de M. Requier, si je partage naturellement l'objectif de cet amendement visant à associer les territoires ultramarins à la gouvernance de l'agence, cette précision nous semble superflue. La notion de « collectivités territoriales et leurs groupements » permet d'ores et déjà de prévoir qu'un représentant des collectivités ultramarines siège au conseil d'administration de l'agence. Il reviendra donc au pouvoir réglementaire de le prévoir, et nous resterons vigilants, bien évidemment, sur ce point.

L'amendement n° 49 de M. Bonhomme vise à apporter une précision supplémentaire dans la composition du conseil d'administration de l'agence. Ce faisant, il me semble ouvrir une brèche qu'il nous sera difficile de refermer ensuite. En effet, si l'on inclut des personnalités qualifiées du secteur de l'ingénierie, pourquoi ne pas également prévoir la présence de personnalités qualifiées oeuvrant dans le secteur de la transition écologique, des professions médicales pour participer à la mission de l'agence concernant l'accès aux soins, des opérateurs pour participer à la mission du numérique, mais également des acteurs du monde des transports ou encore de la revitalisation des territoires ? C'est donc une demande de retrait. Quel est l'avis

d'une agence nationale de la cohésion des territoires, les représentants des territoires soient majoritaires au conseil d'administration. C'est tout ! Cela ne remet nullement en cause le rôle de l'État, puisque, je le répète, le directeur général sera nommé par l'État. Ce refus catégorique de votre part nous inquiète beaucoup.

vote. Je vais m'inscrire dans le droit fil de ce que vient de dire ma collègue Sophie Primas. Je suis moi aussi particulièrement étonné de la position qui vient d'être prise par Mme la Ministre, puisque,

oui ! Manifestement, tout est fait pour que les collectivités ne soient pas présentes ou, en tout cas, ne soient pas en mesure

Nous avons beaucoup de respect pour tous les représentants de l'État. Il y a des personnes de qualité partout, notamment parmi les serviteurs de l'État, mais il ne faut pas non plus se retrouver dans un système technique, voire technocratique, dans lequel les élus de proximité ne sont pas entendus.

vous n'avez pas le contrepoids des élus locaux pour garantir que c'est une vision beaucoup plus équilibrée, et pas simplement budgétaire et financière, qui prévaut,

que l'agence ait un statut et un fonctionnement un peu différents, avec un délégué général et un directoire, ainsi qu'un conseil de surveillance, dans lequel les élus

Alors, je vous le dis, avec beaucoup de respect pour la personne que vous êtes et pour la fonction que vous occupez, si vous voulez réformer en profondeur ce pays, vous ne pourrez pas le faire, ni vous, ni le Premier ministre, ni son gouvernement, ni le Président de la République, sans rétablir la confiance avec les élus locaux. C'est ce que tous ici nous avons exprimé dans le respect des uns et des autres ! Parce que c'est un problème de confiance qui est en cause,

de tous les territoires, notamment ruraux, au sein du conseil d'administration de l'agence. L'objectif est d'éviter une surreprésentation de certains territoires.

et prévoit que ce rattachement peut s'effectuer dès lors que son conseil d'administration l'approuve aux deux tiers de ses membres. Nous souhaitons supprimer cet article pour trois raisons : d'abord, la disposition introduite évoque une notion de rattachement qui n'est pas suffisamment établie sur le plan juridique ; ensuite, le « rattachement » de tels établissements nécessiterait des modifications législatives particulières au-delà de la seule demande des deux tiers des membres de leur conseil d'administration enfin et surtout, il convient que l'État puisse, au-delà des délibérations prises par le conseil d'administration de ces établissements, se prononcer expressément sur

posée. Aller jusqu'à permettre à des agences de décider elles-mêmes, sans que le Parlement en ait décidé, de fusionner avec cette agence de la cohésion des territoires, franchement, les bras m'en tombent

Guillaume Gontard. Par cet amendement, nous revenons sur la structuration de cette agence. Au-delà de sa représentation nationale et des conventions qui seront passées avec d'autres opérateurs, le préfet de département serait donc l'unique représentant territorial de cette agence. On pourrait considérer que cette représentation est naturelle, tenant au fait que le préfet représente l'État. Pour autant, cette représentation unique interroge et interpelle quant à ses conséquences sur les autres acteurs locaux. Ainsi, des représentations territoriales des opérateurs partenaires que sont l'ANRU et l'ANAH ? Le préfet aura-t-il la main sur ces représentations et sur leur financement ? également des autres représentations départementales des services déconcentrés de l'État ? Le choix laissé au seul préfet de département de déterminer, parmi les financements et les différents projets des collectivités, ceux qui relèvent des crédits de l'État sur différents budgets de programme ou du budget de l'agence ou d'autres établissements publics de l'État, porte atteinte à la fois au principe d'autonomie fonctionnelle des établissements publics vis-à-vis de l'État, mais aussi à l'organisation des pouvoirs publics, notamment eu égard aux responsabilités spécifiques des préfets de région dans l'exécution des crédits des programmes dans le cadre des lois de finances. On assiste avec cette représentation préfectorale à la volonté, non pas d'une décentralisation renforcée comme vous l'énonciez, madame la ministre, mais, à l'inverse, d'un fonctionnement très vertical, autour d'un pivot ultra puissant, point unique d'entrée pour les collectivités. Nous sommes très inquiets de cette concentration des pouvoirs au sein d'une seule personne, qui deviendrait ainsi omnipotente et omnisciente, reprenant la main sur l'ensemble des financements en direction des collectivités.

Compte tenu de l'objectif d'un guichet unique pour les collectivités territoriales et du rôle similaire déjà reconnu au préfet de département pour la mise en oeuvre des actions de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, la commission, qui a jugé important de maintenir cette organisation, a émis un avis défavorable.

est à M. Stéphane Artano. La commission du développement durable a procédé à la création de comités de la cohésion territoriale dans chaque département, comités chargés du suivi des projets soutenus par l'ANCT. Ces comités réuniront les représentants des collectivités territoriales et les autres acteurs locaux, qu'ils soient publics ou privés. Si cette intention est hautement louable, nous considérons qu'il revient à l'agence d'assurer un tel suivi. La mise en oeuvre d'une plateforme informatique pourrait remplir cette fonction afin de permettre à ceux qui le souhaitent, y compris les citoyens, d'être informés de l'ensemble des projets en cours dans tous les territoires et de faire émerger des retours d'expériences. Il pourrait également être utile d'y recenser l'ensemble des compétences disponibles localement. Quant au recours à ces comités, nous estimons que cela ajoutera de la complexité et créera une charge de travail supplémentaire qui sera accomplie, nous dit-on, sans aucun frais, ce dont nous doutons. Le suivi des projets de l'ANCT, qui peuvent être très nombreux sur les territoires, demande un véritable investissement en termes de moyens et de temps. Nous pensons que les élus sont suffisamment sollicités. D'ailleurs, comment déterminera-t-on les représentants des élus et des acteurs publics ou privés ? Enfin, ces comités relèvent non des règles constitutives de l'établissement public mais plutôt du pouvoir réglementaire. Le présent amendement vise donc à supprimer

Nous avons soutenu la création proposée par la commission d'un comité de la cohésion territoriale réunissant l'ensemble des acteurs locaux pour le suivi de l'exécution des projets soutenus par l'agence.

Nous espérons que ce comité aura réellement les moyens de fonctionner, qu'il se réunira régulièrement et qu'il ne s'agira pas d'une énième commission Théodule dans laquelle la voix des élus ne compte bien Par cet amendement, nous souhaitons préciser plus particulièrement que les services de l'État intéressés dans le département soient associés aux travaux de ce comité territorial. En effet, comme nous l'avons déjà dit, nous considérons que la création de l'agence de la cohésion des territoires n'épuise pas la compétence de l'État en la matière. Les services déconcentrés de l'État, et non pas le seul préfet de département, doivent donc rester des interlocuteurs privilégiés pour les élus locaux. Je pense notamment à la direction départementale des territoires, à la direction ou encore à une représentation départementale de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Le but de la rédaction proposée pour l'article 5 par la commission n'est pas de créer une structure lourde, contraignante et inutile. Il s'agit de répondre à la demande des élus locaux d'être associés au suivi des actions de l'agence au plus près du terrain. Cette structure locale est politique au sens noble du terme. Elle complète utilement la structure technique nationale

Il permettra à chaque collectivité territoriale de suivre la répartition des soutiens humains et financiers accordés par l'agence aux projets locaux et de veiller à ce que l'action de l'agence ne lèse aucun territoire. La commission a donc émis un avis favorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

: La parole est à M. Mathieu Darnaud. Cet amendement vise à associer les parlementaires et les collectivités locales aux décisions de l'agence. Il convient de créer dans chaque département une commission dont l'avis sera consultatif pour les subventions inférieures ou égales à 100 000 euros et obligatoire au-delà.

mais à construire, à partir du souhait exprimé par les collectivités, des projets pour leurs territoires. L'objet de cet amendement, à savoir une meilleure association des élus locaux à l'action territoriale de l'agence, nous a semblé satisfait par la rédaction introduite en commission à l'article 5 avec la mention du comité local de la cohésion territoriale. Néanmoins, madame la ministre, dans le cas où l'État déciderait de retirer la DETR aux élus locaux pour l'affecter à l'agence, il conviendrait de prévoir la mise en place d'une commission sur le même modèle que celle qui est

par le conseil départemental ou le conseil régional ! Ce serait s'immiscer dans le rôle des financeurs que sont les collectivités locales ou l'État ! Telle n'est pas la vocation de l'agence nationale de la cohésion des territoires.

que les financeurs se mettent autour de la table. De plus en plus, les préfets appellent les collectivités pour savoir si elles financeront ou pas les projets,

des services aux communes. Une coopération entre ces agences départementales et le délégué de l'agence nationale de la cohésion des territoires me paraît de nature à améliorer l'efficacité de l'ingénierie publique sur un périmètre équivalent à celui du

Gontard, sur l'article. Cet article traite des ressources de la future agence. Le moins que l'on puisse dire, c'est que, pour l'instant, celles-ci sont particulièrement floues. Madame la ministre, vous avez répondu lors de votre audition la semaine passée qu'il s'agissait simplement d'additionner les subsides des différents opérateurs intégrés. Or, nous le savons tous, si nous souhaitons que cette agence acquière la force de frappe nécessaire et qu'elle réponde réellement à ses missions, il lui faut beaucoup plus. D'ailleurs, le Conseil d'État partageait cette analyse dans l'avis qu'il a rendu la semaine passée. Nous regrettons à ce titre qu'aucun fléchage n'ait pu nous être indiqué sur un budget prévisionnel de l'agence au titre du projet de loi de finances pour 2019. Nous sommes également inquiets en matière de personnes, puisque la masse salariale des agences est toujours revue à la baisse, dans une trajectoire qui souhaite limiter le nombre de fonctionnaires en poste. Par ailleurs, subsistent des incertitudes sur les modalités de fonctionnement de cette agence. Aurons-nous affaire à un prestataire qui fait payer ses interventions, à l'image du CEREMA et de l'EPARECA, ou s'agira-t-il d'un opérateur aux missions d'intérêt général agissant gratuitement auprès des collectivités ? Ces incertitudes entachent la bonne compréhension de votre projet et font peser des doutes sur la nature même de ce nouvel opérateur. Nous souhaitons, pour notre part, que les prestations de l'agence, ou plutôt ses missions, soient exercées à titre gratuit dans une logique de service publique plutôt que dans une logique marchande dont souffrent déjà beaucoup trop les services publics. Le risque alors serait que seules les collectivités ayant les moyens puissent faire appel à cette nouvelle structure.

Nous l'affirmons, telle n'est pas l'intention du groupe du RDSE, puisque, dans le cadre de la présente proposition de loi, nous n'entendons pas créer de charge supplémentaire pour les collectivités territoriales ni préparer un désengagement de l'État. Bien au contraire, comme nous l'avons rappelé à maintes reprises lors de la discussion générale, il s'agit d'aider en priorité les territoires qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour accomplir leurs projets. Par le présent amendement, nous proposons de préciser que les prestations de service susceptibles d'être facturées sont celles qui correspondent aux missions de l'EPARECA, conformément au droit en vigueur.

La seule exception à ce principe, je l'ai précisé et M. le rapporteur l'a rappelé, est celle qui porte actuellement sur les missions industrielles et commerciales de l'EPARECA et qui donnent lieu à facturation. C'est déjà le cas actuellement, puisque l'EPARECA est un établissement public industriel et commercial. En dehors de cette exception, qui existe déjà aujourd'hui et qui continuera à exister demain, l'appui de l'ANCT ne donnera lieu à aucune facturation

n° 35 rectifié. Nous ne souhaitons pas que la future agence nationale de la cohésion des territoires soit habilitée par la loi à créer des filiales, sans autre précision. Nous estimons que cette possibilité est contraire à la volonté affichée par les promoteurs de cette agence de lisibilité et de clarification de l'action publique. Fusionner différents opérateurs au sein de l'agence pour ensuite filialiser les différentes activités, ce n'est ni cohérent ni le gage d'une efficacité renforcée. De manière plus pernicieuse, nous craignons, par ce biais, la mise en place d'une privatisation rampante et par tranche des services de l'État et de ses opérateurs. Il n'est en effet nullement spécifié que ces filiales devront être totalement ou majoritairement publiques. Voilà une privatisation qui se ferait utilement sans avis du Parlement et donc sans débat. une privatisation qui pourrait apparaître comme une solution utile alors que l'argent public se fait rare et est utilisé pour des dispositifs fiscaux au profit des plus riches, à l'image du CICE. Ce serait aussi une solution convergente et compatible avec la politique de réduction de l'action publique, renforcée par les conclusions du CAP 2022. À l'aune du contexte de création de cette agence, nous voyons très bien les risques sans contrôle et sans filet de cette filialisation. C'est la raison pour

Cet amendement vise à supprimer la représentation des ARS au sein du comité d'action territoriale. Le comité d'action territoriale, qui constitue autour du directeur général de l'ANCT le lieu d'échange, de coordination, entre l'agence et les opérateurs non intégrés, a fait l'objet d'un certain nombre de modifications par votre commission. Parmi ces modifications, l'alinéa 7 prévoit que le comité d'action territoriale comprend des représentants des agences régionales de santé. Outre le fait que les ARS ne disposent pas d'instances de représentation distinctes, le Gouvernement estime qu'elles n'ont pas vocation à intégrer ce comité d'action territoriale, outils d'animation et de coordination de l'ANCT et des opérateurs avec lesquels il a passé des conventions prévues à cet article 7. De surcroît, surcroît, le comité d'action territoriale est composé de représentants des opérateurs de l'État. Il ne serait pas cohérent d'y adjoindre des représentants de services déconcentrés. En effet, les agences régionales de santé ne sont pas des opérateurs de l'État, mais sont des services déconcentrés qui relèvent du ministère des solidarités et de la santé. Si l'on comprend la démarche ayant conduit à intégrer les ARS dans le comité d'action territoriale, cette modalité de représentation du ministère de la santé au sein de l'agence n'est pas adaptée. Par conséquent, le Gouvernement souhaite supprimer la présence

l'avis de la commission ? Sur le fond, je me félicite que les notions de renforcement territorial de l'accès aux soins et de l'offre de soins soient incluses dans les missions de l'agence, car ce sont des éléments fondamentaux de la cohésion territoriale, au même titre que le numérique ou les mobilités. mobilités. Les motifs juridiques avancés par le Gouvernement pour revenir sur la présence de représentants des directeurs généraux des agences régionales de santé au sein du comité d'action territoriale de l'ANCT peuvent être discutés. Il existe ainsi un collège des directeurs généraux des agences régionales de santé, témoignant du fait que les ARS sont structurées « verticalement ». Madame la ministre, au même titre que la téléphonie mobile

Mme Maryse Carrère. La proposition de loi initiale précisait que les conventions conclues entre l'agence nationale de la cohésion des territoires et les établissements publics intervenant dans des domaines connexes ou complémentaires déterminent les conditions de participation et de financement de ces derniers. Le Conseil d'État l'a souligné dans son avis sur la proposition de loi, « ces conventions constituent des modalités essentielles de la coordination de l'action des autres services et opérateurs de l'État que l'agence devra assurer ». Conformément aux objectifs de la création de l'ANCT, et afin qu'il existe une cohérence dans la mise en oeuvre de la politique d'aménagement du territoire par l'ensemble des opérateurs qui interviennent en la matière, le présent amendement tend à faire apparaître les conditions de participation et de financement dans ces conventions. dans ces conventions. Quel est l'avis de la commission ? L'objet de telles conventions conclues entre des établissements publics et l'État est précisément de définir dans quelle mesure et selon quelles modalités ces établissements participent au financement et à la mise en oeuvre de projets communs.

au moment où il faut trouver des équilibres budgétaires ! M. Dallier a raison de dire qu'en l'état de la gravité de la situation et des besoins de la politique de la ville, nous devons impérativement en tant que législateurs sanctuariser l'argent de l'ANRU consacré à ces politiques. à ces politiques. En effet, même si des efforts ont été faits, les sommes actuelles ne sont pas à la hauteur des besoins, qui sont considérables. Je sais bien comment, petit à petit, au nom d'un partenariat ou d'un cas particulier,

nous, renforcer le rôle du Parlement. La commission considère que l'information du Parlement doit être renforcée, en lien avec sa mission constitutionnelle de contrôle et d'évaluation de

en partie aux problématiques soulevées par M. Dallier, mais de manière plus globale. Les conseils d'administration des différents établissements publics de l'État impliqués auprès de l'agence nationale de la cohésion des territoires doivent, non pas avoir simplement connaissance des conventions passées avec l'agence, mais bien valider les conventions pluriannuelles établies entre l'État, l'agence nationale de la cohésion des territoires et les établissements publics. Cette validation semble nécessaire dès lors que ces conventions ne seront pas sans conséquences- c'est le moins qu'on puisse dire -sur les travaux de ces établissements publics, lesquels se trouveront engagés très lourdement auprès de l'agence.

de lenteur, voire de blocage, de l'action de l'agence. Si la concertation entre ces établissements publics est bien le but recherché dans la proposition de loi, il ne faudrait pas en alourdir les modalités. L'avis est donc défavorable.

Guillaume Gontard. Il s'agit d'un amendement de précision. Nous souhaitons affirmer que les futurs fonctionnaires de l'ANCT seront bien en position normale d'activité, et non pas en détachement. Si, pour les fonctionnaires de l'État actuellement en fonction et en position de détachement, des dispositions assurent bien la poursuite du détachement au sein de la nouvelle agence, le recrutement des fonctionnaires doit se faire en position normale d'activité, comme le veut la règle en vigueur pour les établissements publics de l'État. la commission ? Cet amendement vise à préciser que l'agence devra compter dans ses rangs uniquement des fonctionnaires en position normale d'activité. Cette disposition nous semble trop restrictive, y compris pour les fonctionnaires qui y seront affectés et dont l'horizon de carrière serait par trop réduit.

nous ne souhaitons pas que cette future agence puisse procéder à l'embauche de salariés de droit privé. En effet, les missions particulières qui lui sont confiées nécessitent le recours exclusif à l'emploi de droit public, comme c'est le cas pour les établissements publics administratifs. L'emploi public est à nos yeux gage d'efficacité, de compétence et de sens du service public. Nous préconisons ainsi que les agents du CGET, de l'Agence du numérique et de l'EPARECA soient repris sous contrat public, comme la loi le permet. Quel est l'avis de la commission ? de la commission ? Le caractère hybride de l'agence, entre établissement public administratif et établissement public industriel et commercial, suppose de prévoir la possibilité qu'elle emploie, à la fois, des fonctionnaires de l'État, des contractuels de droit public et des salariés de droit privé. Au-delà, ce mélange entre différents statuts d'emploi doit constituer un enrichissement pour l'agence et lui permettre d'exercer au mieux ses missions. À titre d'exemple, l'Agence du numérique est aujourd'hui composée à 80 %, voire à 90 % de salariés de droit privé, et l'EPARECA emploie 43 salariés de droit privé. Dans ces conditions, comment pourraient-ils être intégrés à l'agence nationale de la cohésion des territoires si celle-ci n'a pas reçu de la loi la faculté d'employer des personnels régis par des statuts différents ? L'avis est donc défavorable, par cohérence avec l'intégration de l'EPARECA et de l'Agence du numérique dans l'ANCT.

Le présent amendement vise à préciser les modalités d'intervention de l'ANCT- maîtrise d'ouvrage ou vente et marchés de travaux -quand elle agira dans ce cadre, à l'instar de l'EPARECA actuellement.

nous verrons comment le texte prospérera à l'Assemblée nationale. Il est évident que de ce point crucial dépendra la suite des choses. Nous sommes satisfaits d'avoir pu exprimer, au travers de l'amendement d'Hervé Marseille, la position qui a

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande